sont prévues deux dispositions s'agissant de ces cotisations sociales : une expérimentation d'auto-liquidation, c'est-à-dire la possibilité pour un travailleur indépendant de déclarer dans l'année ses revenus et de payer automatiquement ses cotisations, et la commande d'un rapport du Gouvernement au Parlement examinant les propositions retenues pour simplifier le calcul de l'assiette des cotisations. Pour une raison que je ne m'explique pas, l'article 16 prévoit une première mesure destinée à simplifier le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, en inscrivant dans le code de la sécurité sociale une formule mathématique censée le simplifier. En deux mots, le problème est le suivant : les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une assiette de revenus dite nette, c'est-à-dire diminuée du montant des cotisations sociales que le travailleur est censé devoir payer.

Je vous invite donc à sous-amender l'amendement que nous proposons. Sur le fond, je ne suis pas certain de la portée juridique du présent amendement. Le téléservice, fondé sur une déclaration de revenus des travailleurs indépendants, n'est qu'un instrument d'aide au calcul et ne peut servir en aucun cas de rescrit social.

indiquée dans la loi, alors qu'elle ne peut actuellement qu'être déduite des différents renvois entre le code de la sécurité sociale et le code général des impôts. Il nos yeux d'offrir une meilleure intelligibilité du mode de calcul. Vous indiquez dans l'exposé des motifs de votre amendement que les taux de cotisations retenus dans la formule de calcul

Vous m'interpellez sur le passage de l'assiette nette à l'assiette brute. Je vous confirme que nous souhaitons travailler dans cette direction et que nous envisageons de changer le mode de calcul dans ce sens, mais seulement à moyen terme. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de l'inscrire dans la loi. Nous pensons donc que la suppression des évolutions rédactionnelles proposée conduirait à maintenir un flou sur les dispositions actuellement en vigueur et à faire perdurer pour les travailleurs indépendants une situation assez inintelligible,

trois quarts des travailleurs indépendants pensent que la réforme est une bonne chose, notamment parce qu'elle s'accompagne d'une meilleure relation avec les cotisants. Je pense à l'expérimentation de la relation personnalisée, qui permet à un travailleur indépendant de joindre facilement un agent en cas de litige sur le montant calculé des cotisations.

Cet amendement vise également à supprimer l'article 17, qui introduit une gradation des sanctions applicables en matière de travail dissimulé. Cet article est révélateur de la volonté de l'État de dérégulation en faveur des entreprises, et s'inscrit à contre-courant des positions adoptées par la Cour des comptes. En effet, dans un rapport de 2014, puis dans celui du 7 février 2018, la Cour insiste sur l'importance de relancer les politiques de lutte contre les fraudes aux cotisations sociales en raison de l'enjeu financier majeur qu'elles représentent. Je rappelle que le travail illégal est non seulement une infraction pénale

Dans ces conditions, le bon sens voudrait que de nouvelles mesures soient prises pour que les contrôles soient plus fréquents et les sanctions, plus systématiques, suivant les recommandations de la Cour des comptes. Pourtant, alors que les mesures visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales sont sans cesse renforcées et que le Gouvernement multiplie les mesures austéritaires visant à diminuer la dette sociale, cet article vient adoucir les sanctions applicables en cas de travail dissimulé. Nous nous interrogeons sur le message qui est ainsi envoyé. Cela donne en effet l'impression qu'il existe deux poids, deux mesures dans la sanction des fraudes, et nous nous y opposons. Les entreprises doivent respecter la loi et être sanctionnées lorsqu'elles ne le font pas, d'autant que, comme la Cour des comptes le rappelle dans son rapport, la fraude aux cotisations sociales présente un élément intentionnel, bien loin de la simple erreur. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 17.

il n'est évidemment pas question d'alléger les sanctions, à des requalifications de relations avec des sous-traitants en contrat de travail, qui, avouez-le, sont d'autant moins graves que le fautif est parfois de bonne foi.

Or la carte de service constitue une disposition conventionnelle concernant un outil professionnel. Le présent amendement de clarification vise à mettre fin à une insécurité et à une instabilité juridiques liées à des interprétations diverses et contradictoires de décisions judiciaires. C'est dans cette logique qu'il convient de modifier l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Quel

à ce que fait la société. Si je comprends bien, vous proposez de supprimer le plafond d'exonération de cotisations et contributions sociales applicables aux avantages tarifaires accordés par les opérateurs de transports publics urbains à leurs salariés. La question n'est pas

monsieur le ministre,

France. Quel est l'avis de la commission ?

L'article 18 prévoit l'ensemble des transferts financiers entre les branches de la sécurité sociale et entre l'État et la sécurité sociale entraînés par les exonérations et diminutions de cotisations sociales. Parmi les mesures prévues dans cet article, je retiens la modification de la destination de la taxe sur les salaires- actuellement destinée aux branches vieillesse,

services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et de 6,6 % de ce produit au financement des établissements accueillant des personnes âgées. La part affectée à la section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie passe de 70,5 % du produit de la CASA à 61,4 %, soit une baisse de 9,1 points, tandis que la part du produit de la CASA affectée aux concours versés aux départements pour les actions de prévention diminue de 4,1 points, pour s'établir à 23,9 %.

au vieillissement prévoyait d'adapter 80 000 logements privés aux contraintes de l'âge et du handicap. Mais, entre 2015 et 2017, seuls 45 000

Enfin, l'article 18 prévoit la revalorisation des petites retraites agricoles dans le plan 2014-2017. Cette disposition me permet de réitérer notre volonté d'une application de notre proposition de loi en faveur d'une retraite agricole minimale à 85 % du SMIC, afin de sortir les retraités agricoles de la précarité. Je

à 500 millions d'euros en 2019, avec une perspective de retour à l'équilibre, à partir de 2020, puis d'excédent. Cette embellie cache toutefois des fragilités sérieuses. Premièrement, les perspectives de retour à l'équilibre sont en fait très corrélées à la conjoncture et, si l'activité économique se révélait, dans les années à venir, moins favorable que prévu, le risque qu'une dette sociale ne se reconstitue serait important. Deuxièmement, si la situation s'améliore, c'est en réalité au prix de contraintes importantes qui pèsent sur les hôpitaux, dont le déficit s'est dramatiquement creusé- il s'élevait à 900 millions d'euros l'année dernière et atteindra probablement entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d'euros cette année.

la fragilité de la situation financière de l'assurance maladie et la soutenabilité sur le long terme de notre système de santé sont de plus en plus préoccupantes, au regard de la transition épidémiologique, qui conjugue un accroissement des maladies chroniques avec le vieillissement de la population.

L'année dernière, le PLFSS comprenait des mesures sur la vaccination, la hausse de la fiscalité sur le tabac, ou encore le dépistage, mesures que nous avons toutes soutenues. En revanche, le PLFSS pour 2019 en est dépourvu. Et nous sommes toujours dans l'attente de mesures fortes sur les enjeux de santé environnementale, dont nous savons l'importance qu'ils sont en train de prendre. réforme, celle du système de soins en faveur d'une prise en charge plus adaptée à la transition épidémiologique, de la réorganisation de l'hôpital, d'un renforcement des complémentarités entre médecine hospitalière et médecine de ville et d'une réflexion sur les parcours, qui

dépourvu. Monsieur le ministre, comment afficher un retour au vert des comptes de la sécurité sociale et transférer les excédents vers le budget de l'État quand l'hôpital va aussi mal et quand les réformes nécessaires pour transformer nos systèmes de santé exigent des investissements qui ne sont pas au rendez-vous ?

Quelle protection sociale pour le XXI siècle ? Quel nouveau paradigme pour la sécurité sociale ? Quatre décisions concourent, à mon sens, non-compensation des pertes de recettes, le remplacement de cotisations sociales par la CSG et la nouvelle trajectoire tracée pour les années 2020 à 2022. Il est

Par ailleurs, l'ONDAM fixe un cadre financier et la négociation conventionnelle entre la CNAM et les organisations professionnelles établit les règles de fonctionnement de la médecine de ville, mais les dispositions prévues pour 2019 me semblent aller beaucoup plus loin. Elles dessinent une double évolution : une interpénétration financière quasi

régi par les décisions annuelles du budget de l'État, le budget de la sécurité sociale devenant, comme les autres budgets, une variable d'ajustement. Vous le savez tous, mes chers collègues, la sécurité sociale, c'est une histoire et une autre ambition. C'est la volonté d'apporter une réponse de qualité aux aux accidents de la vie, dont le plus menaçant est, certainement, la maladie. C'est la volonté de construire cette réponse sur des critères qui ne sont

assurées par des dispositions fiscales. C'est un glissement insidieux auquel nous assistons. J'en prends pour preuve deux éléments ponctuels- on pourrait en citer d'autres : la volonté du Gouvernement

irresponsabilité accrue de nos citoyens, soit débattu par le Parlement et fasse l'objet d'une réflexion dans le cadre de la réforme constitutionnelle.

on est en droit de se dire qu'il existe un véritable gisement d'économies. Encore faudrait-il amorcer des réformes de structure. Certaines me paraissent déjà engagées ; je pense en particulier, puisque j'évoque les actes inutiles ou redondants, au dossier médical partagé, le fameux DMP,

pour tirer les conséquences des multiples exonérations et abaissements de cotisations sociales patronales que nous n'avons pas cessé de dénoncer. Par exemple, il prévoit la perte de 22,6 milliards d'euros pour la branche maladie du régime général, qui est compensée par l'État le transfert d'une partie des recettes de la TVA. Quand on sait que la TVA est l'impôt le plus injuste pour nos concitoyennes et nos concitoyens, le transfert de ses recettes vers la sécurité sociale est un moyen supplémentaire de justifier le maintien de taxes, sous prétexte qu'elles sont indispensables, notamment au financement des hôpitaux. Surtout, l'article 19

pleuvent au nom de l'emploi, alors que chacun sait qu'elles ont prouvé leur inefficacité en la matière. Je rappelle avec force que la sécurité sociale doit garantir à chacune et à chacun le même niveau élevé de droits. Ce n'est pas ce que vous proposez avec le présent projet

sur un sujet sur lequel nous voulons montrer notre détermination. L'article 19, nous le comprenons bien, est au coeur de ce que le Gouvernement s'évertue à appeler la rénovation des relations financières entre la sécurité sociale et l'État, soit l'institutionnalisation du principe des vases communicants entre les comptes de la sécurité sociale et le budget de l'État, soit encore la mise sous tutelle de la santé des Français C'est la fin de l'autonomie budgétaire de la sécurité sociale, qui avait été sanctuarisée, entre autres, par la loi Veil de 1994. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous vous êtes appuyés dès la discussion générale sur les exceptions qui ont eu cours par le passé en matière de non-compensation.

par les cotisations sociales vers l'impôt. L'objectif prioritaire est la recherche d'économies aux dépens du modèle social. Tout se tient pour dessiner les contours d'une protection sociale du XXI siècle, qui a été annoncée par le Président de la République et qui serait donc largement rétrécie. Votre conception de la protection sociale, nous le craignons, consiste en un basculement vers un système d'assistance universelle. Mais universalité ne doit pas vouloir dire baisse de la qualité : une prise en charge minimale par les pouvoirs publics et à compléter, si tant est que l'on en a les moyens, par des assurances complémentaires privées, généralisées à tous les pans de la protection, ce n'est pas notre conception de l'organisation de la protection sociale du XXI siècle. C'est pourquoi nous demandons la suppression

qu'il doit rester un outil permettant aux sachants de décider, et non décider à la place de ceux qui doivent le faire, c'est-à-dire le Parlement et le peuple. Cela me paraît évident.

il a aussi voulu le suffrage universel du Président de la République ! La parole est à M. Pascal Savoldelli,

et réalisent des profits- c'est le but d'un patron, pour être très clair -et ceux qui produisent de la force, de la valeur ajoutée et contribuent, aussi, à la croissance et à notre économie ? C'est un débat de société

Nous proposons donc, avec cet amendement, de revenir sur le remplacement des élections aux caisses de la sécurité sociale par la désignation des organisations syndicales et patronales. Cette proposition est un retour à la modernité d'un système fondé sur la démocratie et sur une gestion partagée des richesses entre les travailleuses et travailleurs, et les employeurs. Nous sommes convaincus que le rétablissement de ces élections ouvrira le débat sur les dépenses de la sécurité sociale et les besoins de financement nouveaux, tout en favorisant le retour d'un sentiment de gérer soi-même ses propres affaires.

principe illustre bien la nécessité de clarifier les relations entre l'État, les assurés et la sécurité sociale. Depuis le 1 octobre, les salariés ne paient plus de contributions d'assurance chômage.

Il s'agit d'un bouleversement majeur, car ce régime était, jusqu'à présent, d'essence assurantielle, à la fois financé par des contributions et versant, en cas de perte d'emploi involontaire, des prestations en fonction de l'ancien salaire, c'est-à-dire des contributions de l'intéressé. Que va devenir ce régime, et que vont devenir ces prestations, une fois que les salariés ne contribueront plus et que l'impôt se substituera à eux ? Ceux-ci seront-ils toujours des assurés, disposant des droits acquis par eux-mêmes à travers des contributions versées par leur employeur ou bien n'auront-ils désormais droit qu'au traitement social que la société voudra bien leur accorder ? Avouez que c'est tout de même une question de fond, monsieur le ministre, et que l'on a réglé le problème sans véritable débat de fond

ce qui se cachait derrière l'assurance chômage. En d'autres termes, d'ici à quelques années, la différence de prestations en fonction du salaire sera-t-elle toujours légitime ? C'est une question ! L'avenir de l'assurance chômage tient-il en une prestation uniforme, sur le modèle du filet de sécurité, financé par l'impôt, que percevront certains indépendants- je rappelle que la somme est modeste : 800 euros par mois

Et c'est bien le chemin que, en toute logique, les partenaires sociaux, qui en discutent actuellement, semblent emprunter.

Pour assurer la neutralité de cette modification, nous proposons une mesure qui nous paraît, d'ailleurs, beaucoup plus logique. Elle consiste en la prise en charge des cotisations salariales par les employeurs, la baisse à due concurrence des cotisations patronales à la branche famille et un fléchage de la CSG destinée à l'UNEDIC

En 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé contraire à la réglementation européenne ce type de prélèvements. Malgré un nouveau fléchage, l'État s'est de nouveau fait condamner en 2018 par la justice administrative française. Pour anticiper une décision non favorable du Conseil d'État, nous étudions aujourd'hui cet article du PLFSS, tendant à supprimer la CRDS et la CSG sur les revenus fonciers encaissés par les Français de l'étranger à l'étranger, quand ils se trouvent dans l'Union européenne, dans l'espace économique européen et en Suisse.

les Français de l'étranger qui vivent en dehors de l'Europe et de la Suisse ont le sentiment qu'il existe une double catégorie de Français : ceux de l'Europe et ceux du reste du monde. Moins bien traités, moins bien considérés, ils vivent cette décision comme une véritable injustice. Or, monsieur le ministre, rien ne vous empêche d'étendre cette exonération à l'ensemble des Français vivant à l'étranger, indépendamment de leur communauté.

la totalité des Français vivant dans le monde de la CRDS et de la CSG sur les revenus fonciers qu'ils encaissent en France. Il tend, d'autre part, à exonérer les non-résidents français du nouveau prélèvement de solidarité de 7,2 % sur les revenus fonciers, ainsi que sur les produits de placement.

Depuis six ans, l'ensemble des représentants des Français de l'étranger ne cessent de répéter que la situation des Français établis hors de France vis-à-vis des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers n'est pas normale. Soumettre une personne à des prélèvements sociaux alors qu'elle ne bénéficie d'aucun régime de sécurité sociale et qu'elle relève d'une autre législation en cette matière est discriminatoire, en plus de heurter le principe d'égalité devant l'impôt.

Vous projetez en effet de supprimer la CSG uniquement pour les personnes résidant dans l'Union européenne, alors que toutes les sommes prélevées entre 2012 et 2015 au titre des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des non-résidents fiscaux français doivent être remboursées, et pas uniquement celles qui les résidents de l'Union européenne. L'objet de cet amendement est donc d'étendre la portée de cette exonération à toutes les personnes relevant de la législation d'un autre État en matière d'assurance maladie et qui ne sont pas soumises à un régime obligatoire de sécurité sociale français au cours de l'année, sans aucune distinction de résidence. Le Gouvernement a choisi de ne pas écouter l'ensemble des représentants des Français établis hors de France qui l'alertaient cependant sur les risques juridiques liés aux prélèvements sociaux. conséquence, 59 000 recours en remboursement ont été introduits contre l'État. Mme Genetet elle-même, qui est issue de votre propre parti, recommande dans son rapport de supprimer les prélèvements sociaux sans distinction du lieu de résidence. Elle qualifie par ailleurs le contentieux lié à ces prélèvements de véritable bombe à retardement. Je vous propose donc de désamorcer cette bombe ! Les

qu'ils louent ; pourquoi les obliger à payer des cotisations sociales alors qu'ils ne bénéficient d'aucun système de sécurité sociale ?

les dispositions qui ont été insérées par l'Assemblée nationale au sein de l'article 19 changent la donne, puisqu'elles répondent rigoureusement au droit communautaire tel qu'il a été énoncé par la Cour de justice. Nous ne nous situons nous situons donc plus sur le terrain du droit européen, mais dans le cadre politique purement français. Que sont la CSG et la CRDS ? Il s'agit d'impositions de toutes natures qui n'ouvrent pas de droits- c'est un point important un point important -, mais se trouvent simplement affectées à la sécurité sociale. Leur objet même est de frapper la quasi-totalité des revenus perçus en France, dans une optique purement contributive. Dès lors, le fait que certains de nos compatriotes acquittent ces contributions sans être inscrits à la sécurité sociale française ne diffère en rien du fait qu'ils aient à acquitter d'autres taxes ou prélèvements destinés au budget de l'État, alors même, par exemple, qu'ils n'empruntent pas les routes nationales ou que leurs enfants ne vont pas à l'école en France. Pour autant, estimerions-nous normal que ces Français ne paient aucun impôt français sur des revenus français ? Je ne le crois pas. Dans cette affaire, la sécurité sociale a simplement constitué un cas particulier pour un nombre limité de personnes inscrites dans un autre régime européen, du seul fait qu'il existe un règlement communautaire spécifique sur ce sujet.

aujourd'hui nous avons progressé dans la transcription, si j'ose dire, de la jurisprudence dans notre législation.

En effet, s'il est légitime que l'État puisse bénéficier, dans une certaine mesure, du retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, ces coupes ne sont pas acceptables en l'état : en premier lieu, parce qu'elles préemptent dès à présent des excédents hypothétiques dont la réalité devra être constatée en deuxième lieu, parce qu'elles ne semblent pas compatibles avec le remboursement de la dette résiduelle de la branche maladie et du FSV d'ici à 2022, selon la trajectoire définie par le Gouvernement lui-même en annexe B ; en troisième lieu, parce qu'il est nécessaire que le Gouvernement et le Parlement s'entendent sur les principes qui régiront l'équilibre à long terme des comptes sociaux, par exemple lors de la réforme institutionnelle à venir ou d'un débat que nous organiserions en ce sens, avant de prendre des mesures jusqu'en 2022. À cet égard, la remise d'un rapport du Gouvernement ne saurait engager à elle seule l'ensemble des pouvoirs publics, même si ce point fondamental est versé au dossier. Il est donc proposé de supprimer les réaffectations de ressources prévues

à la fois fiscalement domiciliés à l'étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français, y compris les adhérents à la Caisse des Français à l'étranger, ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS dont nous avons parlé, au moins au titre de leurs pensions.

à la CFE, ou à un système équivalent, qui couvre la prise en charge de soins des Français de l'étranger quand ils se trouvent à l'étranger. Cette double imposition dont le montant total représente environ 8 % est aujourd'hui due par l'ensemble des retraités français vivant à l'étranger, quel que soit le montant de leur retraite. Elle est évidemment lourde pour les non-résidents fiscaux percevant une « petite retraite » quand il s'agit de leur seule pension.

exonérer de la COTAM les Français de l'étranger retraités qui encaissent tous les mois une somme inférieure à 900 euros. Il

en cas d'arrêt maladie, leur salaire maintenu par la sécurité sociale après trois jours de carence. Toutefois, comme dans de nombreux secteurs d'activité, la convention collective garantit un maintien de salaire dès le premier jour d'arrêt maladie.

reprises par la Cour des comptes. La présente mesure vise à rendre effective l'application d'un jour de carence pour les agents des organismes de sécurité sociale, dans le prolongement de la décision d'instaurer un jour de carence dans la fonction publique. Il s'agit d'une mesure d'équité entre agents publics, d'autant plus justifiée que, dans un certain nombre d'organismes comme les agences régionales de santé, et agents de droit privé d'organismes de sécurité sociale. Cette mesure renforcera également l'efficience des organismes de sécurité sociale, leur permettant d'atteindre les objectifs de réduction des coûts de fonctionnement, sans pour autant remettre en cause le service rendu aux assurés sociaux. sociaux. Quel est l'avis de la commission ?